sur la défense. Dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l’auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répartie pendant une minute.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, évoquer les questions de défense en Europe était iconoclaste. En dehors des préoccupations en matière d’élargissement, de marché unique, de zone euro et d’accords commerciaux, point de salut ! Aujourd’hui, les Européens sont rattrapés par une réalité violente. Face à nous, des États ont tout misé sur la puissance, considérant que les traités et principes internationaux sont des barrières de papier. Je le rappelle, trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU ont adopté des comportements problématiques. Dès 2008, la Russie a mené une guerre éclair en Géorgie, puis s’est attaquée à l’Ukraine en 2014 et 2022. La Chine se dote rapidement de tous les moyens économiques, technologiques et militaires pour bouleverser l’ordre mondial à son profit. l’attitude des États Unis inquiète. Donald Trump a accéléré le processus de divergence entre les partenaires transatlantiques et se concentre sur ses objectifs : la Chine et l’Iran. Son obsession pour l’Arctique le conduit à vouloir mettre la main sur le Groenland. Pour défendre ses intérêts globaux, le président américain semble disposé à sacrifier l’Ukraine, et peut être la sécurité de l’Europe. mais les États membres ne se posent pas tous la question de la défense dans les mêmes termes. La plupart considèrent que la défense de l’Europe relève de l’Otan et du parapluie nucléaire américain, d’où leurs faibles investissements nationaux.

Ce changement d’approche et d’échelle implique une mobilisation rapide qui semble optimiste, au regard notamment de la complexité des sujets, du nombre de domaines capacitaires identifiés comme prioritaires et de l’ampleur des efforts à conduire pour faciliter la mobilité militaire. La mobilisation de moyens financiers extraordinaires est impérative. La Commission évoque un plan de 800 milliards d’euros qui correspond essentiellement à de la dette des États, voire à de la dette commune. Il ne faudrait pas que ces mécanismes deviennent un moyen de contrôle par Bruxelles de la défense des États membres. Le livre blanc rappelle aussi la nécessité d’encourager les financements privés au profit des entreprises de défense, en particulier des PME. C’est la reconnaissance d’un problème longtemps occulté. Pour suivre le sujet depuis plusieurs années, je connais les difficultés pratiques rencontrées par de nombreuses entreprises et je ne suis pas certain que toutes les réticences des acteurs financiers soient durablement levées. Les défis industriels et économiques sont immenses pour produire des volumes importants, à moindre coût, tout en sécurisant et en diversifiant les filières d’approvisionnement. La future politique de stocks sera, elle aussi, très coûteuse. Si l’accroissement des dépenses militaires se confirme, il doit se faire au profit des entreprises européennes, dans un cadre de coopération renforcée.

rien de précis n’est dit concernant la préférence communautaire. L’expérience montre que certaines acquisitions ont été faites à l’étranger en dépit de l’existence de solutions européennes équivalentes et compétitives. C’est évidemment troublant, et il ne faut pas s’imaginer que les Américains vont abandonner le marché européen, alors qu’un afflux de crédits est imminent. Et je ne parle pas de la Corée du Sud d’Israël. Les questions de concurrence intracommunautaire et les règles d’exportations hors Union européenne ne sont pas non plus à négliger. en général les initiatives de la Commission, et de son actuelle présidente, avec une certaine prudence. Sa propension à se mêler de tout, à interpréter avantageusement les traités et à surréglementer est avérée. La Commission est aussi à l’origine de la taxonomie européenne, dont le classement conduit à ne pas reconnaître comme durables les activités liées à la défense, quand les concurrents étrangers bénéficient, eux, d’un large soutien public et privé. Il faudra voir comment, sur la taxonomie et d’autres contraintes européennes, les choses évoluent concrètement puisque des simplifications sont annoncées. Je note que peu de développements sont consacrés au Royaume Uni. Quelle sera sa place exacte ? En dehors de la France, c’est la seule autre puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité,

C’est un premier pas concluant, une initiative bilatérale qui pourrait servir de modèle à une plus grande échelle. Les États Unis laisseront ils les autorités britanniques jouer un rôle comme elles l’entendent ? Néanmoins, ce réveil est tout de même le signe positif d’une prise de conscience des enjeux de sécurité en Europe. Il faudra veiller à préparer la guerre de demain probablement une guerre de haute intensité, mais peut être aussi une multiplication d’actions indirectes et multichamps, en « zone grise », sous le seuil de conflictualité, donc difficiles à attribuer, auxquelles il est plus compliqué de répondre.

opérationnels, nous défaire des lourdeurs administratives, porter une attention particulière à la chaîne de sous traitance, mais également renforcer les ressources humaines, militaires et industrielles, sans lesquelles rien ne sera possible. Je note que déjà certains industriels européens font venir de la main d’œuvre d’Asie. Pour conclure, nous sommes clairement à un tournant de l’Histoire.

Je vous remercie, Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ces dernières semaines, des négociations se sont tenues en Arabie saoudite entre l’Ukraine, les États Unis et la Russie, sans l’Union européenne.

Rappelons quelques faits. À l’automne 2021, plusieurs mois avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Pologne, mais aussi la Lituanie, pays résolument tournés vers le camp occidental et attachés à l’Union européenne, sont victimes d’une attaque hybride menée par la Russie et la Biélorussie. le principe ? Exercer une pression migratoire ingérable à leurs frontières. L’Europe s’est mobilisée, notamment avec Frontex, mais certainement pas suffisamment. Pourquoi ? Parce que les fondements mêmes de l’Union européenne ont été ceux d’une union économique. Ils ont été ceux d’une union pour la paix par la prospérité et non, pour reprendre les mots d’Ursula von der Leyen au sujet de l’Ukraine, de la paix par la force. Les bouleversements géopolitiques de ces dernières années nous obligent à changer d’approche.

La guerre en Ukraine a ensuite donné lieu à de nombreuses initiatives, comme la boussole stratégique et une redéfinition du rôle de l’Union européenne sur la scène internationale. La réélection de Donald Trump à la tête des États Unis, son rapprochement avec la Russie et sa décision de suspendre les aides américaines à l’Ukraine nous obligent à aller plus loin. C’est dans ce contexte que la Commission européenne a dévoilé en mars dernier le très attendu livre blanc sur la défense européenne. Si l’Otan reste la pierre angulaire de la défense collective de l’Europe, l’Union a désormais le devoir d’assurer sa propre sécurité. Le soutien à l’industrie européenne de la défense est un point majeur de ce livre blanc. Partant du constat que trop peu d’initiatives communes européennes voient le jour en ce domaine, la Commission européenne a identifié plusieurs secteurs critiques dans lesquels des projets réunissant au moins deux pays européens doivent être menés. Tel est par exemple le cas de la défense aérienne et antimissile, ou encore de l’intelligence artificielle. Afin de mieux préparer l’Europe aux scénarios les plus pessimistes, la Commission européenne préconise d’améliorer les mobilités militaires en constituant des stocks et en renforçant nos frontières extérieures, notamment avec la Russie et la Biélorussie. Enfin, le soutien à l’Ukraine est au cœur de ce livre blanc, qui prévoit une assistance militaire accrue et une plus grande intégration des industries de défense européenne et ukrainienne. Ces mesures s’accompagnent bien évidemment de propositions financières financières ambitieuses. C’est tout le sens du plan ReArm Europe, qui a été présenté par la Commission européenne au début du mois de mars et validé sur le principe par l’ensemble des États membres lors du Conseil européen du 6 mars dernier. Les dispositifs proposés dans ce plan visent à mobiliser jusqu’à 800 milliards d’euros pour notre défense. Le plan prévoit notamment une dérogation au pacte de stabilité et de croissance qui permettra aux États membres de dépenser davantage pour leur défense sans être visés par une procédure de déficit public excessif. Afin de financer les

Je rappelle que lors des Conseils européens des 6 et 20 mars dernier, les vingt sept États membres ne sont pas parvenus à un consensus sur l’Ukraine à cause de la Hongrie. Demain, il est possible que d’autres États membres bloquent les décisions. N’oublions pas que pendant des années, les États membres se sont divisés sur les questions de défense,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un nouveau livre blanc de la défense était nécessaire ; il était attendu depuis longtemps. Il était nécessaire, parce que le contexte géopolitique a profondément changé depuis 2022, date de la parution de la feuille de route dite boussole stratégique. également nécessaire parce que nous devons impérativement prendre le virage d’une véritable défense européenne. Ce document très attendu, aurait dû tracer les grandes lignes d’une politique commune pour les années à venir et promouvoir une indispensable autonomie stratégique, est au fond décevant.

Plus précisément, ce livre blanc manque de portée et de cohérence. Le document propose des mécanismes pour améliorer la coopération et la coordination interétatiques en vue d’un marché unique, mais il ne prévoit aucune structure claire et incitative visant à faire converger les actions politiques des États. La mutualisation des budgets de défense des États pour des acquisitions conjointes, fer de lance du programme Edip (), n’est pas mentionnée. Manquent également des solutions de financement novatrices et communes. Le document propose certes un investissement colossal de 800 milliards d’euros, mais, dans les faits, 150 milliards d’euros seraient à la charge des États, sans prise en compte de leur capacité d’endettement nationale. Pour les 650 milliards d’euros restants, aucune réelle solution de financement n’a été avancée. La seule option financière nouvelle est la possibilité, pour les États membres, de renoncer à la TVA dans le cadre de l’instrument Safe, ce qui représenterait des montants ridiculement faibles. Il aurait fallu aller plus loin, en envisageant par exemple la défiscalisation totale de l’ensemble des filières de production de la défense. Une solution sérieuse consisterait notamment à modifier la taxonomie européenne afin de permettre au système financier de soutenir l’industrie de la défense. À ces deux écueils majeurs, j’ajouterai deux critiques encore plus problématiques, car révélatrices des options philosophiques qui sous tendent notre défense européenne. La première le réarmement européen ne vient qu’en réaction au conflit russo ukrainien et que le cadre stratégique proposé a pour vocation première d’intégrer l’Ukraine dans l’architecture de sécurité européenne, en l’associant aux initiatives de l’Union,

faire de l’Alliance atlantique, et donc, en creux, des États Unis le centre de gravité géostratégique de la défense européenne me paraît être une grave erreur, notamment en raison de l’imprévisibilité de la politique américaine. Le livre blanc aurait dû proposer clairement un repositionnement des responsabilités entre l’Union européenne et les États membres. La vocation de l’Union européenne est d’organiser efficacement le marché unique de la défense. Les États membres, eux, doivent assurer la gestion des personnels et des opérations militaires au travers, par exemple, d’une alliance entre les États disposant déjà de capacités militaires opérationnelles, en y incluant notamment le Royaume Uni et la Norvège.

nous sommes réunis ce soir pour débattre du livre blanc de la Commission européenne sur la défense. Je remercie le groupe Les Républicains de cette initiative utile. Avant d’aller plus loin, permettez moi de déplorer vivement, amèrement, qu’un tel document,

ce que ce livre blanc n’est pas. Il n’est pas un document fixant une chimérique stratégie supranationale de défense européenne. Il n’est pas, non plus, une feuille de route qui poserait les bases d’une armée européenne intégrée.

Et pour être tout aussi clair, rappelons que notre politique de défense repose sur les piliers fondamentaux que sont la revue nationale stratégique, qui a pris la suite des livres blancs, une loi de programmation militaire (LPM) et des lois de finances qui, chaque année, traduisent les ambitions Ce triptyque existe et continuera d’exister. Après avoir évoqué ce que n’était pas ce livre blanc, j’en viens donc à ce qu’il est. Il constitue tout d’abord une reconnaissance des positions que la France porte avec constance depuis de nombreuses années. Dès septembre 2017 – le président Patriat s’en souvient –, dans son premier discours de la Sorbonne, le Président de la République affirmait qu’au fondement de la communauté politique est la sécurité. « Nous vivons en Europe […] un désengagement progressif et inéluctable des États Unis », précisant immédiatement qu’« en matière de défense, notre objectif doit être la capacité d’action autonome de l’Europe, en complément de l’Otan ». Que d’énergie a t il fallu déployer pour faire accepter à tous les États européens ce qui paraît aujourd’hui une trivialité, une lapalissade, une évidence : le concept d’autonomie stratégique européenne, qui a été gravé dans le marbre de la boussole stratégique européenne durant la présidence française de l’Union, en 2022 Ce livre blanc, qui accompagne le plan ReArm de l’Union européenne, est aussi une validation du choix effectué par la France en 2017, et même

Le réveil est brutal pour ceux qui avaient mis tous leurs œufs dans le même panier transatlantique, moquant la volonté française d’autonomie européenne comme un ersatz de gaullisme suranné, dans ces années 2000 qui fleuraient bon la fin de l’Histoire. Mais le retour au réel est là. La guerre durable en Ukraine a fait prendre conscience de la dépendance sécuritaire en matière de renseignement, du caractère désormais imprévisible de l’allié américain, qui suspend l’aide américaine à l’Ukraine, mais donne des cartouches à Vladimir Poutine pour différer tout cessez le feu véritable.

menacent de diviser nos sociétés à coups d’infox et d’influence, sapant la cohésion nationale comme européenne. Dans ce contexte, le livre blanc est un bon début

l’Union européenne face à un monde qui devient compétitif, face aux menaces et aux interrogations qui pèsent sur l’avenir de la garantie de sécurité américaine. Avant d’ailleurs

En vingt ans, la part de l’Europe dans les dépenses militaires mondiales est passée de 27 % à moins de 16 %. Dans le même temps, la part de la Chine a doublé. La Russie, malgré un appareil productif fragilisé, consacre encore plus de 6 % de son PIB à la défense. Pendant ce temps, l’Europe a réduit ses arsenaux, sous investi dans ses capacités et parié sur l’attraction des dividendes de la paix. Depuis que la Russie constitue une menace existentielle pour l’Europe, la réalité est limpide. La compétition entre puissances ne se cache plus derrière les traités. La Russie transforme le champ de bataille de l’Ukraine en laboratoire d’une guerre d’attrition. La Chine étend patiemment ses réseaux logistiques, de l’Indo Pacifique à la Méditerranée. Et les États Unis, désormais dirigés par une administration désignée par Donald Trump, lequel assume une lecture purement transactionnelle des alliances, nous rappellent que l’article 5 du traité de Washington n’est plus une promesse inconditionnelle. Dans ce contexte, la France, seule puissance nucléaire de l’Union, a évidemment un rôle à jouer. Sans renier l’indépendance de la doctrine nucléaire, elle peut contribuer à la sécurité des Européens par une concertation stratégique approfondie. Nos intérêts vitaux ont une dimension européenne. Il est donc légitime que nos partenaires soient associés à une réflexion sur les conditions dans lesquelles notre dissuasion contribue à la stabilité du continent. Cette réflexion commune n’équivaut ni à un partage ni à une délégation ; elle constitue la marque d’une responsabilité et d’une confiance sans faille à l’égard de la souveraineté européenne.

La clause dérogatoire du pacte de stabilité permettra aux États membres d’augmenter temporairement leurs dépenses militaires jusqu’à 1,5 % du PIB. Si ce levier est indispensable, sa mise en œuvre doit s’inscrire dans le cadre d’un suivi solide, afin d’éviter que cette clause ne serve qu’à requalifier des dépenses déjà budgétisées. Dans cet esprit, il nous semble que la création de l’instrument Safe, qui autorise la Commission à lever 150 milliards d’euros sur les marchés pour financer les investissements de défense, est le plus ambitieux des mécanismes du livre blanc. Le groupe du RDSE qu’il plaide depuis longtemps pour un emprunt européen commun au service de l’autonomie stratégique. Le principe de cette dette mutualisée pour financer les achats conjoints est une avancée politique majeure que nos partenaires européens des pays dits frugaux commencent à entendre. entendre. Le livre blanc de la défense propose enfin de mobiliser l’épargne privée la Banque européenne d’investissement. Cette stratégie ne nous semble pas immédiatement pertinente eu égard à la préservation du modèle social qui est Avant de solliciter l’épargne des Françaises et des Français, il serait judicieux d’explorer les mécanismes de contribution des entreprises les plus aisées, en premier lieu celles du secteur de la défense, qui bénéficieraient directement de ces investissements.

Nous saluons enfin les mesures en faveur de l’Ukraine, notamment l’intégration de son industrie dans les chaînes européennes. Cette solidarité ne doit toutefois pas masquer l’essentiel : nous devons préparer l’Europe aux scénarios de haute intensité.

Ce livre blanc ne doit donc pas en rester au stade de la déclaration d’intention. Il doit déboucher sur une programmation claire, cohérente et suivie. Le groupe du RDSE soutiendra tous les instruments budgétaires et industriels qui permettront d’ancrer cette dynamique dans les politiques publiques des États. La parole

Elle est peuplée par 450 millions d’habitants et dotée d’un PIB de 18 000 milliards d’euros, ce qui en fait la deuxième économie mondiale. Les pays européens dominent les classements de développement humain, nos écoles attirent le monde entier et nos cultures influencent bien au delà de nos frontières. l’Union européenne a tout d’une grande puissance, n’ayant rien à envier à ses grands compétiteurs internationaux. Néanmoins, s’il est un domaine dans lequel cette grande puissance reste un colosse aux pieds d’argile, c’est la défense. Depuis 1945, les États européens ont privilégié la protection des États Unis, pays allié, mais lointain, plutôt que d’investir dans leur propre défense, sans pour autant considérer leur éventuel retrait. Le général de Gaulle disait : « Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts. » C’est aussi vrai pour l’allié américain. Aujourd’hui, les yeux de Washington sont rivés sur le Pacifique et la Chine, alors que l’isolationnisme américain ressurgit violemment. Outre Atlantique, on s’interroge : « Pourquoi mourir pour l’Europe ? Nos dollars doivent ils financer la défense des Européens ? » L’actuel président américain semble avoir tranché. Le constat pour l’Europe est sévère : nous avons accumulé un trop grand retard dans nos politiques militaires et nous ne sommes pas en mesure de faire face aux menaces qui nous entourent. La France a depuis longtemps fait le choix d’une autonomie stratégique, se dotant de l’arme nucléaire et d’une armée complète pouvant être déployée partout autour du monde. Cependant, elle ne peut concourir dans la course à l’armement que les superpuissances américaines, chinoises ou russes se livrent. Nos nombreuses tentatives pour structurer une politique de défense commune au sein de l’Union sont longtemps restées lettre morte, nos partenaires européens privilégiant la protection américaine. Pourtant, le constat du renforcement et de l’autonomisation nécessaires de nos forces armées semble aujourd’hui faire consensus. Si les Européens veulent la paix, ils doivent désormais se préparer à la guerre. Ce réveil brutal de la guerre en Europe, nous aurions dû l’anticiper dès le 24 février 2022, avec la violation russe du territoire ukrainien, au mépris de toute légalité internationale. Qui peut croire que la Russie s’arrêtera à l’Ukraine, alors qu’elle renforce massivement son armée, sa marine et son industrie d’armement ? Qui peut croire que le dictateur du Kremlin n’attaquera pas l’Europe si elle est faible et délaissée par les États Unis ? Qui peut croire qu’abandonner nos alliés ukrainiens au sort que leur réserve Vladimir Poutine garantira la paix sur notre continent ? Restons éveillés : la Russie s’arme contre nous et les États Unis préparent dans notre dos les conditions d’une paix inacceptable pour l’Ukraine, dont nous ferons inévitablement les frais. Si nous voulons nous protéger, mais aussi protéger nos valeurs, nos idées, nos acquis sociaux et sociétaux, l’ensemble des vingt sept membres de l’Union européenne doivent mener une politique de réarmement, de Lisbonne à Tallinn, de Stockholm à Athènes. Soulignons les initiatives de nos partenaires européens, notamment l’Allemagne, qui planifie d’ores et déjà des investissements massifs pour la défense. Ces efforts salutaires outre Rhin sont décisifs pour accompagner et soutenir le mouvement collectif de renforcement militaire. Cependant, ce réarmement européen ne sera pas immédiat, tant le retard est grand. La majorité des armées européennes se sont structurées comme des forces de soutien à l’armée américaine, non comme des forces de projection indépendantes. La dotation matérielle de ces mêmes armées dépend de la BITD américaine. Enfin, notre coordination stratégique doit être renforcée, prenant acte des forces et des faiblesses des armées de chaque État membre. Le livre blanc pour la défense, publié le 19 mars 2025 par la Commission européenne, apporte une réponse à ces nombreux défis à l’horizon de 2030. Pour financer la préparation stratégique des États membres, l’Union européenne se dotera d’un nouvel instrument appelé Sécurité et action pour l’Europe (Safe), correspondant à des prêts garantis par le budget de l’Union à hauteur de 150 milliards d’euros sur quatre ans pour les investissements militaires et technologiques des États membres. Par ailleurs, comme lors de la crise du covid 19, l’Union activera la clause de sauvegarde du pacte de stabilité et de croissance pour une hausse équivalant à 1,5 % du PIB du budget de la défense de chaque État membre. Cette souplesse permettrait une croissance sur quatre ans d’environ 650 milliards d’euros pour les investissements dans la défense. Au total, 800 milliards d’euros d’investissements pour la préparation de la défense seraient donc projetés sur quatre ans. Ce livre blanc cible aussi les priorités européennes pour notre résilience stratégique : les armes aériennes, aéroportées, l’artillerie, les stocks de munitions, les drones, la logistique, l’innovation technologique et la protection des infrastructures. Veillons néanmoins à ce que ces armes soient bien fabriquées sur notre sol, tout en respectant la souveraineté des États. La Commission entend renforcer ses liens stratégiques avec le Royaume Uni, la Norvège, le Canada, la Turquie, mais aussi auprès des États voisins de l’Union, ainsi qu’auprès de ses partenaires dans l’Indo Pacifique, tout en rappelant que la stratégie de défense européenne ne peut se passer de l’Otan, pierre angulaire de notre coordination. Enfin, elle précise que les relations avec les États Unis doivent être entretenues, mais conscientes. Les intérêts américains ne convergent pas et ne convergeront pas toujours avec les nôtres. La question du Groenland en est un parfait exemple, et les forces militaires des États de l’Union européenne doivent être en mesure de dissuader les ambitions expansionnistes du 47 président des États Unis. Dans un monde qui se réchauffe, d’un point de vue non seulement climatique, mais aussi géopolitique, les Européens doivent redoubler d’efforts pour se doter d’une force militaire multiple, apte à dissuader comme à opérer, résiliente et capable de défendre nos intérêts et nos valeurs. Avec la chute de l’Union soviétique et la domination incontestée des États Unis, nous, Européens, avons cru naïvement à la fin de l’Histoire. Nous avons cru en un monde de paix sous la protection du gendarme américain, où nous pourrions devenir les rentiers des dividendes de la paix. Nous y avons cru et nous avions tort. Les jours de paix se couchent à l’ouest ; la nuit tombe à l’est, entraînant avec elle son lot de guerres et d’incertitudes. Spectateurs de ce sinistre crépuscule, nous devons unanimement pour une meilleure coordination stratégique, industrielle et logistique de notre défense. Ensemble, nous sommes plus forts. C’est pourquoi le livre blanc pour la préparation de la défense publié par la Commission européenne est un pas en avant historique pour dissuader nos adversaires, sans oublier le réarmement moral qu’il nous faudra conduire. La

visent à renforcer le pilier européen de l’Otan et à renforcer l’interopérabilité de nos armements avec ceux qui sont définis par l’Otan. D’ailleurs, les domaines capacitaires qui sont inclus dans le livre blanc correspondent peu ou prou à ceux qui avaient été identifiés par l’Alliance. sur le plan politique, vous l’avez rappelé, se posent des questions quant à la garantie de sécurité américaine et à la posture des États Unis au sein de l’Otan, en particulier au moment où l’on voit les

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes amenés, à l’occasion de la publication de ce livre blanc, à débattre de la stratégie globale de l’Union européenne en matière de défense. Ce document traduit un aveuglement et une incompréhension sur les causes des conflits actuels. Pis, la Commission européenne ne tire pas les leçons du passé. Le bilan de trente ans d’élargissement de l’Otan vers l’Est et la nécessité d’une évolution des discussions sur notre sécurité collective en Europe sont ignorés, alors que notre continent s’enfonce dans l’escalade des tensions avec notre voisin russe. De même, la plupart des Européens considèrent qu’ils n’ont autre choix que de continuer la guerre, alors que l’objectif doit être une paix négociée, qui ne soit pas une capitulation de l’Ukraine. Nous sommes contraints de constater, mes chers collègues, après trois années de conflit, que la stratégie guerrière laisse derrière elle un bilan dramatique de morts et de sacrifices. Alors que, au printemps 2022, à Istanbul, Kiev accepte la neutralité et que, en contrepartie, Moscou concède un retrait de ses troupes des territoires occupés depuis février 2022, les pays occidentaux les plus préoccupés par le cas de Poutine ont préféré livrer des armes à l’Ukraine, plutôt que de répondre favorablement aux garanties de sécurité demandées par celle ci. En induisant Kiev en erreur avec la livraison d’armes, cette stratégie présente un risque. À l’occasion d’un accord de paix ressemblant davantage à un accord de capitulation, ces armes pourraient tomber dans les mains d’un régime ukrainien revanchard et souhaitant reconquérir par la force les territoires perdus, perdus, avec le risque de déclencher à terme un nouveau conflit régional. Le livre blanc souhaite avancer vers l’Europe puissance, mais ce document mal conçu se confronte à des contradictions. Le chapitre sur nos partenariats stratégiques en est la preuve. L’Union européenne souhaite un renforcement des coopérations en accord avec nos valeurs, mais se vautre dans des inadmissibles Turquie d’Erdogan, qui enferme le maire d’Istanbul, ou avec l’Inde de Modi, qui multiplie les actes discriminatoires et autoritaires dans son pays. Enfin, parler de « situation fragile » à Gaza, comme le font les auteurs de ce livre blanc, c’est méconnaître ou, pis, ignorer le génocide commis au mépris du droit international et reconnu par l’ONU. Ce « deux poids deux mesures » dans nos condamnations participe de l’effondrement du droit international et renforce l’envie de nos adversaires de le contourner. Aussi, ce double standard est une manière pour Poutine d’utiliser nos incohérences et de continuer son œuvre funeste avec l’opinion derrière lui, alors qu’il faut détacher la société russe de son emprise. En réalité, derrière ces valeurs progressistes se cache le grand retour de l’idéologie atlantiste. La Commission estime que, pour reconstruire la défense européenne, une étroite collaboration avec l’Otan est nécessaire, ajoutant même que la course aux armements permettrait d’accéder à une autonomie stratégique européenne. Laissez moi douter, monsieur le ministre, face face à une Allemagne, une Pologne et un Royaume Uni projetant d’acheter des missiles et avions américains pour des milliards d’euros au détriment de l’industrie européenne… Cette référence répétée à l’Otan permet surtout d’accorder des Européens divisés en fixant le cap depuis Washington. La France est forcée de marcher au pas. Pourtant, et vous le savez, les États Unis de Trump et Vance, par leurs actes hostiles, ne sont plus nos alliés. Même sans les États Unis, l’Europe surpasse la Russie dans presque tous les domaines. Les États membres de l’Union dépensent déjà 460 milliards La motivation de ces 800 milliards d’euros supplémentaires répond donc à un impératif non pas sécuritaire, mais idéologique. Alors que le secteur automobile européen est en difficulté et que l’Allemagne entre en récession pour la troisième année consécutive, l’ère du réarmement d’après Mme von der Leyen apparaît comme la solution solution miracle. Nous disons non à cette politique de surarmement, qui nous précipite vers l’escalade avec la Russie plutôt que vers la paix. Utiliser la situation actuelle pour perpétuer des rivalités économiques et militaires dans ce contexte n’est pas responsable. Nous appelons à reprendre la voie de la diplomatie et à réaffirmer de la France, comme nous réclamons la restauration des moyens de notre diplomatie. Nous ne pouvons pas donner à notre jeunesse la guerre comme seul horizon, alors que les défis sociaux et environnementaux se multiplient. Ce choix politique de surarmement entraînerait surtout

Enfin, mes chers collègues, j’attire votre attention sur la méthode : notre Parlement n’a jamais pu se prononcer sur les projets de la Commission européenne, qui n’a aucune légitimité démocratique ni compétence en la matière, alors que nous sommes, dans cet hémicycle, élus au suffrage universel, avec la confiance des citoyens et des territoires. Votre chemin n’est décidément pas le nôtre. Si nous voulons la paix, alors préparons la paix, une paix juste et un avenir serein pour nos enfants ! le ministre délégué. Madame la sénatrice Gréaume, quelle inversion des valeurs et quelle inversion des responsabilités ! On ne préparera pas la paix par la soumission,

sur le terrain avec des frappes régulières contre les villes ukrainiennes et maintient des objectifs maximalistes, comme la neutralisation de l’Ukraine, sa démilitarisation, le renversement du président Zelensky… C’est l’effacement de l’Ukraine en tant que nation indépendante que vise la Russie. C’est nous qui sommes ciblés par l’escalade et les menaces permanentes de la Russie avec ses sabotages, ses attaques cyber, ses ingérences, ses menaces contre la souveraineté et les frontières des États européens souverains depuis la fin de la guerre froide. Alors, ne confondons pas les responsabilités, ne nous autoflagellons pas ! Oui, l’Europe sera toujours du côté de la paix et de la liberté, mais, pour défendre la paix, il faut être capable de défendre nos intérêts et il faut être capable de dissuader l’agresseur.

Alors que le recours à l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exclut le Parlement européen de tout droit de regard, ce que nous déplorons évidemment, il est important et bienvenu de pouvoir tenir ici un débat démocratique. Dans les grandes lignes, nous approuvons l’effort engagé par l’Union européenne et ses membres pour démultiplier notre soutien à l’Ukraine et construire les conditions d’une réelle autonomie stratégique continentale. Dans le détail, nous formulerons commentaires, réserves et propositions. Avec 650 milliards d’euros de dépenses à la seule charge des États membres, le plan Réarmer l’Europe laissait à penser que nous allions vers davantage de défense de l’Europe, certes, mais pas vers davantage d’Europe de la défense. Si le livre blanc ne bouscule pas ces équilibres, en raison d’une trajectoire budgétaire européenne trop rigide jusqu’en 2027, il apporte quelques éléments intéressants. Ainsi, le programme Safe prévoit 150 milliards d’euros levés par l’Union européenne sous forme d’emprunts mutualisés, qui ne pourront être décaissés que pour effectuer des achats groupés entre plusieurs pays et auprès de notre industrie européenne de défense, puisque 65 % des crédits devront être consommés pour l’achat de produits ou de composants européens. Monsieur le ministre, nous voyons toute l’influence de la France dans la fixation de cette ambition. Me référant à notre débat lors de l’examen du budget, je me satisfais de cette jauge, qui est ambitieuse, sans être trop rigide, vu l’urgence du contexte et l’ampleur du progrès à accomplir. Nous saluons également l’ouverture de ce mécanisme à l’Ukraine, qu’il s’agisse de la mutualisation des achats entre l’Ukraine et des pays de l’Union ou de la possibilité de comptabiliser la BITD ukrainienne avec celle de l’Union. Compte tenu de la montée en puissance de cette dernière, depuis une décennie, cette évolution est tout à fait bienvenue. Nous croyons cette disposition à même de faire évoluer dans le bon sens des habitudes nationales très ancrées et d’avancer collectivement vers un réflexe essentiel : acheter européen quand une solution européenne existe. Nous notons la tentative de définir des besoins capacitaires et des priorités d’investissement européens. C’est un premier pas, qu’il faudra articuler avec la définition trop souvent autocentrée des besoins nationaux. En ce sens, je n’ai pas le sentiment que le travail de réactualisation de notre revue nationale stratégique intègre suffisamment cette dimension des besoins collectifs de l’Union. J’espère une inflexion en ce sens dans la mouture finale que le Gouvernement présentera avant l’été. un mot sur l’intelligence artificielle et les drones autonomes mentionnés par le livre blanc, car certaines tournures de phrase nous inquiètent. Nous tenons à rappeler ici notre opposition totale à toute évolution de la législation européenne en matière de drones, dans la mesure où celle ci interdit l’utilisation de toute arme autonome capable de tuer un être humain sans décision explicite d’un autre être humain. Dans la même logique, nous appelons l’Union à se doter d’une législation relative à l’utilisation de l’intelligence artificielle, incluant particulièrement ses utilisations militaires. concerne les mécanismes de financement de cet effort considérable, nous restons sur notre faim, quand nous ne sommes pas inquiets. En attendant des financements directs à partir de 2027 dans le prochain cadre budgétaire pluriannuel, nous sommes pour le moment contraints de recourir à l’emprunt, donc à la dette, dette collective et dette de chaque État, permise grâce à un assouplissement temporaire du pacte de stabilité. Cet assouplissement pour les seules dépenses de défense est insuffisant. Il faut réformer intégralement le pacte de stabilité et y inclure les dépenses essentielles des États : la défense, la transition écologique, la justice sociale, les investissements d’avenir. Nous demandons également des investissements européens dans tous ces domaines stratégiques. Nous le répéterons systématiquement : les dépenses militaires ne doivent pas entrer en concurrence avec nos autres dépenses essentielles. L’autonomie stratégique européenne n’existera pas sans transition ni sobriété énergétiques pour arrêter notre dépendance aux énergies fossiles et à l’uranium russe. Elle n’existera pas non plus si des populations paupérisées par l’affaiblissement de nos filets de protection sociale placent l’extrême droite alliée de Poutine au pouvoir. À l’échelle européenne, comme à l’échelle nationale, pour financer notre effort militaire, il faut des ressources complémentaires et de la justice. Ainsi, il est inenvisageable que ces milliards d’euros d’argent public enrichissent éhontément les actionnaires des industries de défense. Il faut encadrer leurs futurs dividendes.

qui sera mis en œuvre dans les prochaines années. Celui ci vise précisément à harmoniser les règles de l’intelligence artificielle sur le marché européen et à susciter des financements et des investissements, tout en encadrant, notamment, son usage sur le plan éthique ou militaire. Vous avez mentionné le cadre financier pluriannuel. Bien sûr, nous défendrons une ambition haute pour le budget de l’Union européenne, en particulier son volet militaire, auquel j’ajouterai le spatial,

pour rattraper notre retard sur nos concurrents, en particulier les États Unis, dans le domaine de la tech, de l’intelligence artificielle, du quantique, de la défense ou encore de la décarbonation.

franchit l’Atlantique pour aller aux États Unis – à hauteur de 300 milliards d’euros par an – de se porter vers nos besoins d’investissement, vers nos start up, vers nos PME. C’est au contraire en faisant de notre continent le plus attractif et le plus compétitif

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il aura fallu les violations du droit international par la Russie, l’arrivée de Trump au pouvoir, son imprévisibilité, ses menaces de désengagement militaire, la mise à l’écart de l’Union européenne des négociations sur l’avenir de l’Ukraine, la multiplication des ingérences dans nos processus démocratiques, pour que l’idée d’une Europe de la défense prenne enfin forme. Nous pensions être à l’abri, jusqu’à ce que le parapluie américain, qui nous protégeait tout en nous vassalisant, menace de se refermer, et nous prenons conscience que l’appartenance à l’Otan n’est plus une garantie de sécurité fiable. Qui peut croire aujourd’hui, après le choc des droits de douane, que M. Trump activera l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord si un pays membre était attaqué ? Après des mois d’alerte sur la nécessité et l’urgence d’une autonomie stratégique européenne, la présentation d’un livre blanc pour la défense est bienvenue. Certes, depuis l’agression de l’Ukraine par M. Poutine, les États membres de l’Union européenne ont réalisé un effort de réarmement sans précédent, mais un effort dans l’urgence, réalisé en ordre dispersé, qui a mis en évidence nos carences, la fragmentation de la BITD européenne, des problèmes d’interopérabilité et, surtout, une dépendance aux importations américaines. Nous vivons un moment de bascule, qui nous oblige à faire preuve de volonté et de courage politique. Nous devons en urgence renforcer nos capacités de dissuasion. L’Europe est riche, développée et stable. Pour reprendre l’expression du commissaire européen à la défense, M. Kubilius, les 450 millions d’Européens ne devraient pas dépendre des 350 millions d’Américains pour se défendre contre 150 millions de Russes. Nous devons assurer notre autonomie, notre défense, notre puissance, et cela passe par une véritable politique coordonnée de défense. Bien qu’il ait été publié tardivement, le plan présenté par la présidente von der Leyen a le mérite d’être lucide sur le contexte géopolitique et démontre une prise de conscience des menaces existantes et de la nécessité d’un réveil européen en ayant pour ambition une autonomie stratégique de l’Europe d’ici à cinq ans. Si de nombreux points quant à la proposition de créer un marché européen de défense sont à discuter et préciser, la volonté de faciliter la circulation des biens de défense au sein de l’Union, d’alléger les charges administratives et le développement de programmes européens conjoints pour certains projets de défense spécifiques sont à souligner. Ce livre blanc n’est qu’une première étape vers l’autonomie que la Commission, il faut le dire, aurait dû franchir bien plus tôt. Ce livre blanc arrive tard, mais il propose aussi trop peu. En effet, nous attendons de la Commission qu’elle joue le rôle de facilitatrice en s’assurant que les États membres investissent prioritairement dans du matériel européen – à cet égard, le plan ReArm Europe et les 150 milliards d’euros de prêt du programme Safe sont bienvenus, mais insuffisants nous avons besoin de beaucoup plus d’argent, et l’on peut regretter les tergiversations des États membres à l’égard d’un emprunt commun de 500 milliards d’euros associé à une préférence européenne. De même, on peut regretter l’absence de consensus pour utiliser les 200 milliards d’euros d’avoirs russes gelés, qui devraient dès à présent permettre à l’Ukraine de résister, de compléter son armement et de préparer sa reconstruction. N’oublions pas que l’Ukraine est notre première ligne de défense et que, dans le face à face américano russe, elle a plus que jamais besoin de la solidarité et de l’aide européennes. Ces financements que nous appelons de nos vœux permettraient par ailleurs de ne pas franchir la ligne rouge de l’utilisation des fonds de cohésion pour financer l’effort de défense. L’exigence d’une sécurité et d’une souveraineté militaire ne peut en aucun cas se faire au détriment de la solidarité territoriale, de nos piliers sociaux et de la lutte pour le climat. Nous ne pourrons pas construire une Europe puissante en fragilisant les territoires et les Européens par plus d’inégalités. Ce livre blanc et ReArm Europe sont une première étape. Ils attestent une volonté et pointent des priorités : dépenser mieux et ensemble pour combler nos lacunes capacitaires, renforcer notre dissuasion grâce aux technologies de rupture, élargir nos partenariats, améliorer la mobilité militaire, agréger les commandes et intégrer la BITD ukrainienne. Tout cela va dans le bon sens, mais il faut accélérer et adopter rapidement le programme Edip, le programme pour l’industrie européenne de défense. Dans le contexte géopolitique actuel, fait de menaces hybrides, ce livre blanc ne peut être la seule stratégie. La réponse aux défis sécuritaires doit nécessairement être globale. La mise en place d’un bouclier démocratique européen en fait aussi partie, pour défendre nos valeurs et la place de l’Europe dans le monde. Nous attendons des dirigeants européens, en particulier de vous, monsieur le ministre, qu’ils prennent leurs responsabilités et apportent une réponse forte et cohérente à la hauteur des enjeux. La parole

déchirer, revenir à des solutions nationalistes et affaiblir la réponse collective de notre continent. Au contraire, nous avons su nous unir et emprunter pour relancer nos économies. Nous faisons face aujourd’hui à un autre moment

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà cinq ans déjà, durant la crise du covid 19, chaque État européen a défendu ses intérêts, quitte à marcher sur son voisin. Puis, la Commission non élue de Bruxelles a contracté des dettes pour relancer l’économie et réindustrialiser. Cinq ans plus tard : toujours rien ! Aujourd’hui, Mme von der Leyen présente un livre blanc pour contracter 810 milliards d’euros de nouvelles dettes dans l’intention de nous réarmer dans les cinq prochaines années. Et nous devrions la croire ? Comme nombre de Français, comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Or tout ce que nous voyons, c’est la dette qui enfle et la pression fiscale qui devient insupportable, sans aucun investissement stratégique à l’horizon ! Les bonnes intentions couchées sur ce papier ne peuvent résister à la réalité. Quand Bruxelles parle de préférence européenne dans la production d’armements, elle n’impose qu’un seuil de 65 % des composants provenant d’Europe, ce qui nous laisse notamment dépendants des procédures Itar (International le livre blanc de Bruxelles ouvre les achats conjoints avec le Royaume Uni, le Canada ou l’Australie, alors que ces derniers nous ont humiliés en annulant le contrat qui devait être historique de douze sous marins nucléaires voilà quatre ans à peine, même s’ils s’en mordent quelque peu les doigts aujourd’hui.

! Vous parlez de souveraineté militaire et de patriotisme ? Vous ne contrôlez même pas les investissements étrangers qui viennent piller ce qui nous reste de vivier industriel ! Et l’on voit aujourd’hui l’entreprise française LMB Aerospace, qui équipe nos hélicoptères, nos Rafales et nos porte avions, passer sous pavillon américain…

Preuve, s’il en est, que la Commission ne parvient toujours pas à concilier les intérêts des Estoniens en même temps que ceux des pays latins ! Bref, quand on parle de réarmer, il nous incombe déjà de pointer du doigt ceux qui ont désarmé. Or, en la matière, nous ne pouvons pas vous faire confiance, à vous qui avez refusé d’entendre le général de Villiers, ni à la Commission européenne, qui s’est construite sur la naïve idée de la fin de l’Histoire et des dividendes de la paix. de la paix. Monsieur le ministre, ne pensez vous pas que nous avons moins besoin d’un livre blanc de la Commission européenne sur la défense que d’un livre bleu blanc rouge pour protéger et développer l’excellente base industrielle de défense française et accorder des moyens à notre armée, qui est et doit rester aux ordres de Paris, et non pas soumise à un conglomérat berlino bruxellois

de naïveté quand vous et vos alliés politiques avez prôné l’alliance avec Vladimir Poutine. Vous avez vous même participé à l’observation électorale des élections truquées en Russie,… Pas plus qu’à Marseille ! … pour légitimer le régime de Vladimir Poutine

même vos alliés politiques le constatent aujourd’hui en Europe : la meilleure réponse face au défi migratoire, c’est évidemment la coopération européenne. C’est évidemment la mise en œuvre du pacte asile et migration, qui permettra

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’Union européenne a dévoilé le 19 mars dernier un document politique majeur, son livre blanc pour une défense européenne, accompagné du plan d’action ReArm Europe. Il s’agit de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union et de soutenir les capacités de défense de ses États membres. Au travers de ce texte, la Commission acte ce que beaucoup d’entre nous constatent ici depuis des années : l’ère des dividendes de la paix est bel et bien révolue ; et, sans base industrielle solide, il ne peut y avoir de puissance stratégique. Face aux nouvelles menaces, à la guerre qui fait rage en Ukraine, à la fragilité croissante de l’ordre international et à la perspective du désengagement américain, l’Europe n’a d’autre choix que de se préparer et de s’armer sans déposséder les États membres de leurs prérogatives régaliennes. Le livre blanc le dit clairement, les investissements européens dans la défense étaient insuffisants, fragmentés et souvent inefficaces. Beaucoup ont nourri le consortium militaro industriel américain, nos voisins et alliés considérant le parapluie états unien comme éternel et hésitant sur les solutions européennes existantes, pour ne pas dire les solutions françaises. L’Europe ne peut plus et ne doit plus confier sa sécurité aux États Unis, un allié qui n’a comme boussole que ses seuls intérêts. L’heure est à la prise de conscience et à la correction, et c’est tant mieux Pour assurer sa propre sécurité, l’Europe ne pourra faire l’économie d’une harmonisation des standards et des procédures, harmonisation qui sera indispensable pour une mise en place efficace d’une interopérabilité entre États membres. Toutefois, dans cette nouvelle ambition européenne, qui passe par le soutien à l’Ukraine ou encore par la consolidation de l’industrie européenne de défense, la France a un rôle central à jouer en tant que puissance nucléaire disposant de compétences reconnues et d’un véritable tissu industriel. Oui, la France est un acteur militaire important au sein de l’Union et au sein de l’Otan. Avec le plan ReArm Europe, la Commission propose plus de 800 milliards d’euros mobilisables répartis autour de trois axes un effort budgétaire national coordonné, la clause dérogatoire du pacte de stabilité ; la création de l’instrument Safe, capable de lever jusqu’à 150 milliards d’euros sur les marchés pour financer des achats conjoints la mobilisation de la Banque européenne d’investissement et de l’épargne privée pour structurer un écosystème industriel de défense pérenne. Ce plan constitue une avancée majeure dans la maturation stratégique de l’Union. Il est à la fois une réponse à l’urgence, en soutenant concrètement l’Ukraine, et une vision de long terme, en favorisant l’innovation et l’autonomie stratégique. Toutefois, permettez moi, mes chers collègues, de formuler trois conditions indispensables à sa réussite. d’abord, l’Europe ne pourra pas se contenter d’un empilement de contributions nationales. Il faudra de la cohérence, de la mutualisation et de la lisibilité budgétaire. Ensuite, le renforcement de notre base industrielle et technologique de défense ne doit pas être sacrifié sur l’autel des achats rapides ou des intérêts particuliers. Le soutien à l’innovation, aux PME et aux capacités critiques doit être central.

sans une volonté politique forte, constante et partagée entre les États membres. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, nation cadre en Europe, a une responsabilité historique dans cette dynamique. Ce livre blanc ne règle pas tout – il ne remplace ni l’Otan ni nos responsabilités nationales –, mais il marque un tournant, un sursaut, une déclaration d’intention forte, celle d’une Europe qui veut non plus subir, mais choisir. La parole

du Pentagone qui est à l’origine d’innovations technologiques comme le GPS ou encore internet – à l’européenne. Renforçons les outils européens dont nous disposons. Je pense par exemple à European Innovation Council, cette agence qui doit investir dans l’innovation en Europe, mais qui pourrait être

a une responsabilité et un rang particuliers à tenir. Elle est une puissance dotée de l’arme nucléaire et un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle défend depuis 2017 l’ambition de l’autonomie stratégique et elle continuera de le faire.

Mouret. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce livre blanc européen, le premier du genre, n’est pas un simple document ; il est l’affirmation d’une volonté politique d’avancer ensemble. Néanmoins, l’ambition ne suffit pas. Encore faut il nous en donner les moyens. Les dépenses de défense des États membres ont, certes, augmenté de 31 % depuis 2021, mais le compte n’y est toujours pas. Si chacun a jusqu’à présent investi selon ses propres priorités, le moment est venu de mutualiser nos efforts. Il est possible de structurer une véritable BITDE grâce à des coopérations industrielles bilatérales ou multilatérales. Je pense à l’accord CaMo (capacité motorisée) avec la Belgique ou au système de défense antiaérienne Mamba avec l’Italie. Mais un obstacle persiste : celui de la concurrence intra européenne entre nos industriels, qui s’ajoute à la concurrence internationale. Monsieur le ministre, n’est ce pas le moment d’envisager un marché intégré ou, en tout cas, de revoir les règles de notre marché intérieur pour aligner nos ambitions stratégiques sur nos pratiques économiques ? Face aux géants qui nous entourent, l’Union est un puissant levier pour faciliter les coopérations, renforcer l’interopérabilité, réduire les coûts, mais aussi soutenir les infrastructures à double usage pour la mobilité militaire et les communications. M. le ministre Lecornu a déclaré que l’argent du contribuable européen ne peut pas être dépensé « pour produire sous licence des équipements américains ». Je partage son point de vue. Il y va en effet de la souveraineté de l’Europe. Cette souveraineté passe d’abord par la réduction de nos dépendances. Où en sommes nous de la désitarisation de nos matériels ? Pourrons nous encore dépendre d’un standard de liaison de données tactiques de l’Otan, alors que des solutions européennes pourraient émerger ? Que faisons nous pour sécuriser nos accès aux matériaux critiques et renforcer une main d’œuvre européenne ? Sur le plan financier, nombre de nouvelles initiatives vont dans le bon sens. Je voudrais néanmoins vous alerter sur la révision du Fonds européen de qu’il subventionne des usines produisant du matériel américain exporté vers les États Unis, comme c’est déjà le cas dans le domaine civil. Ce livre blanc nous invite à penser l’après, un avenir sous la forme d’une alliance européenne étendue au Royaume Uni et à la Norvège, fondée sur l’acquis otanien articulée autour des forces de dissuasion franco britanniques, des moyens terrestres allemands et polonais et des capacités navales espagnoles, grecques ou italiennes. Dans ce paysage, la France peut être le moteur de la défense européenne, du fait non seulement de son modèle de son modèle d’armée complet, de l’excellence de son industrie, mais surtout de sa dissuasion nucléaire entièrement indépendante, potentielle clé de voûte de la sécurité du continent, à condition de prendre des engagements politiques et stratégiques plus fermes. Cela signifie aussi prendre des mesures concrètes et tangibles avec nos partenaires. Monsieur le ministre, au delà des missions de réassurance de l’Otan, n’est il pas temps d’adosser notre garantie de sécurité au déploiement de troupes et de capacités, par exemple en Pologne ? Nos lacunes restent nombreuses en matière de commandement, de défense solaire, de renseignement satellitaire, de frappe dans la profondeur ou encore de guerre électronique. Les combler exigera des investissements colossaux pour soutenir l’Ukraine aujourd’hui et assurer notre sécurité demain. Ces enjeux dépassent les capacités d’un seul pays. Ce livre blanc devra donc irriguer nos politiques nationales. Ces conclusions seront elles intégrées dans la prochaine Revue nationale stratégique, en lien avec les stratégies de défense de nos partenaires ? Monsieur le ministre, de retour d’un déplacement à Washington, je peux vous affirmer que les Américains s’organisent. Ils sont prêts à produire et à exporter pour renforcer leur industrie et créer des emplois chez eux. Et nous, Européens, quel est notre cap ? La parole

d’entendre des engagements fermes de la part du Gouvernement sur les coopérations renforcées que nous pouvons avoir avec nos partenaires. Je pense notamment à la question qui est, je crois, la plus politique,

Belrhiti. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui d’une question cruciale pour l’avenir de la sécurité et de la souveraineté de l’Europe : le livre blanc de la Commission européenne sur la défense. la défense. Ce document présente des pistes pour renforcer les capacités militaires européennes et coordonner la défense sur notre continent. Cependant, il est essentiel de garder à l’esprit que la défense reste une compétence régalienne des États. Nous partageons l’idée qu’une Europe de la défense plus forte est nécessaire, mais nous avons des réserves sur certaines propositions. Nous ne remettons pas en cause la nécessité d’un renforcement des capacités de défense au sein de l’Union européenne, mais nous estimons que ce renforcement ne doit pas signifier la dilution de la souveraineté des États membres. La défense, la gestion des forces armées et la sécurité doivent relever du contrôle des autorités nationales. La Commission européenne doit se limiter à un rôle de soutien et de coordination, sans interférer dans les choix stratégiques de chaque pays. Cela dit, ce livre blanc soulève des enjeux importants pour l’avenir de l’industrie de défense européenne. Nous devons garantir à l’Europe une capacité d’innovation et de production militaire autonome, indépendamment des fournisseurs étrangers. Il est inconcevable que 80 % des dépenses européennes en matière de défense soient encore allouées à des équipements produits en dehors de l’Union, comme le soulignent les auteurs du rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie de 2023. Cette situation expose l’Europe à des dépendances stratégiques dangereuses. De plus, nous appelons de nos vœux l’introduction de critères de préférence européenne dans les actes d’achat de matériel et défense, afin de soutenir prioritairement nos entreprises et technologies locales. Il s’agit non pas d’un protectionnisme à outrance, mais d’une mesure pragmatique visant à garantir l’autonomie stratégique de l’Europe. Si nous voulons une Europe forte, il est impératif que notre industrie de défense soit renforcée et compétitive sur la scène mondiale. Cependant, la coopération avec nos alliés, en particulier au sein de l’Otan, reste un axe stratégique fondamental. L’Europe doit pouvoir agir en coordination avec ses partenaires, mais il est essentiel de ne pas confondre cette coopération avec une intégration supranationale. Chaque État membre doit garder le contrôle sur ses décisions en matière de sécurité. Pour conclure, nous soutenons une Europe de la défense forte et compétitive, mais il est impératif que cette Europe ne se transforme pas en une Union imposant une vision uniforme de la défense. La défense doit rester sous le contrôle exclusif de chaque pays, afin d’assurer une Europe autonome, forte et respectueuse de ses États souverains. La parole

tente, par ses ingérences, d’allumer des contre feux pour promouvoir l’instabilité et le chaos directement à nos frontières ! Nous commémorerons cette année les 30 ans du génocide de Srebrenica et des accords de Dayton Paris, qui ont mis fin à la situation en Bosnie. Si j’évoque ce déplacement, c’est parce qu’il est d’usage d’entendre dans le débat public que la guerre serait de retour sur notre continent depuis le 24 février 2022 et l’invasion de la Russie en Ukraine. Mais la vérité est que nous, Européens, avons été dans une forme de déni de la guerre et de la violence pendant des décennies. La guerre n’avait pas disparu du continent pendant des décennies, mais notre Europe était divisée par le rideau de fer avec des dizaines de millions de citoyens sous oppression soviétique et communiste, cet « Occident kidnappé », comme l’appelait Milan Kundera, derrière le rideau de fer. Puis, dans les années 1990, il y a eu ce que nous avons cru être des anachronismes, le retour de vieilles haines, la guerre dans les Balkans, où nous avons dû attendre l’arrivée des États Unis pour pouvoir mettre fin à un génocide sur notre sol. En 2008, ce fut l’agression de la Russie contre la Géorgie. En 2014, à la suite du mouvement démocratique pro européen du Maïdan, ce fut l’attaque de la Russie contre le Donbass et l’annexion de la Crimée. Et, bien entendu, il y a eu la guerre contre l’Ukraine, avec la menace que fait porter la Russie sur l’ensemble de nos démocraties par ses ingérences, ses sabotages, ses attaques cyber, ses menaces, ses remises en question des frontières et des souverainetés des États libres issus de la fin de la guerre froide. À cela

à ce défi, face à ce retour des conflictualités et des rivalités géopolitiques, faisons le choix de l’union de notre continent. Faisons le choix du réarmement et de la défense collective de nos intérêts, de nos valeurs et de notre sécurité. La parole

Les tensions et les conflits se multiplient dans le monde. La guerre, avec le conflit ukrainien, est aux portes de l’Europe, tandis que les alliances nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont questionnées. Plus que jamais, la question de la défense commune européenne est d’actualité. Mais pour avancer, encore faut il poser le problème dans des termes clairs et sortir du concept général pour préciser le mode opératoire. La première question à se poser est de savoir si l’on parle l’Europe de la défense, laissant à penser qu’il s’agit d’une action communautaire, ou de la défense de l’Europe, ce qui renvoie à une union d’États qui se reconnaissent comme constituant un ensemble ayant des intérêts communs en raison de leur histoire, de leurs valeurs et de leur géographie. Dans le premier cas, il s’agit d’aller vers une Europe fédérale, dans le second, de construire une Europe des États ; rien de bien nouveau, en quelque sorte, depuis le débat sur la Communauté européenne de défense… Le livre blanc ne répond pas formellement à cette question, mais, très clairement, la Commission se propose d’aider les États à identifier les insuffisances et priorités capacitaires, sans préciser d’ailleurs par rapport à quels objectifs précis, ou encore à faciliter l’efficacité, l’interchangeabilité et l’interopérabilité. Or, en l’état des traités, mes chers collègues, je suis désolé de le dire, la Commission n’a formellement ni mandat, ni compétence, ni légitimité pour mettre en place une politique européenne de la défense, donc pour pointer des insuffisances, édicter des priorités ou définir des normes. Il est à noter d’ailleurs que c’est par le prisme de ses prérogatives dans le domaine de la politique industrielle que la Commission tente de fédérer des initiatives autour des industries de défense, en laissant croire qu’il existerait une BITD européenne, ce qui est un abus de langage. C’est un abus de langage, parce que non seulement l’industrie de la défense – vous l’avez dit, monsieur le ministre – ne s’inscrit pas dans une logique de marché et de libre concurrence, aussi parce que ses clients sont les États, au travers des états majors, et que, à ce jour, il n’y a pas d’État européen. C’est sans doute là que se situent les limites du projet Edip, qui peut apparaître, à bien des égards, avant tout comme un outil au service d’une politique industrielle, plutôt que comme une réponse militaire, capacitaire et opérationnelle à l’urgence du moment. En période de tension, l’heure n’est sans doute pas au montage de coopérations industrielles entre plusieurs pays, en espérant des retombées économiques pour chacun d’eux, mais davantage à la désignation de chefs de file

qui devront être approuvés par la Commission, selon des procédures dont la Commission a le secret et dont les principales caractéristiques de fonctionnement ne sont ni la simplicité ni la réactivité. Si nous voulons mettre en place

Le deuxième point que je souhaite soulever est bien sûr celui du financement. Il y a trois mois, on ne parlait que de la dette publique de 3 300 milliards d’euros. Depuis un mois, on n’en parle plus,

qui concerne la France, chacun sait que nous avons déjà explosé tous les compteurs. Augmenter les dépenses pour la défense est sans doute indispensable, mais peut on accroître encore le déficit ? Poser la question, c’est déjà y répondre. Commençons déjà par payer nos fournisseurs, alors que nous avons 8 milliards d’euros de reports de charge. C’est l’un des préalables à la montée en puissance de leur production. Essayons aussi de respecter la loi et les financements qui y sont attachés. Selon des responsables que j’ai récemment auditionnés, le programme 146, « Équipement des forces », aurait été amputé de près d’un milliard d’euros En conclusion, nous ne pouvons qu’approuver une initiative commune aux pays européens pour organiser leur défense. Il y a urgence et nécessité. Sachons transformer une crise en une chance pour bâtir un projet commun. Pour autant, notre réponse ne peut pas se faire dans un cadre opérationnel, juridique et institutionnel approximatif et instable. Le moment est venu de répondre aux questions de fond : où se prennent les décisions, sous quelles formes et avec quelles procédures La France est le seul pays de l’Union à disposer à la fois de l’arme nucléaire, d’une armée de projection et d’une véritable BITD, même si elle ne couvre pas tous les champs des besoins. Cela nous confère des responsabilités, mais aussi une force pour faire valoir nos intérêts. Sachons nous montrer à la hauteur de nos ambitions